La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue, Alain Pluchet, qui fut sénateur de l'Eure de 1983 à 1998.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Cohésion des territoires » (et articles 54 et 54 ).

mais ces crédits restent en baisse de 1,5 milliard d'euros par rapport à la totalité de ceux ouverts cette année, au fil des lois de finances rectificatives. Les dépenses fiscales atteignent 10,1 milliards d'euros, ce qui montre l'importance des dépenses extrabudgétaires pour les politiques de cette mission. S'agissant du programme 177, qui finance la politique d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, il bénéficie de 2,2 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation significative de 209 millions Notons toutefois que ces crédits sont inférieurs à ceux inscrits en cours d'année 2020, car la crise sanitaire a conduit le Gouvernement à ouvrir 450 millions d'euros supplémentaires. Cette rallonge a permis d'assurer jusqu'à présent une gestion correcte de la situation, hormis le triste incident de l'évacuation du camp de Saint-Denis, une opération massive de mise à l'abri mobilisant 34 000 places d'hébergement supplémentaires, dont 12 000 nuitées hôtelières. L'un des enjeux de 2021 sera donc, avec des moyens en baisse, d'assurer l'accompagnement et la transition des personnes vers des centres d'hébergement, puis vers un logement pérenne.

que l'année 2020 a connu un nouvel exercice de régulation budgétaire avec la révision soudaine, le 14 juillet dernier, des critères de subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour l'isolation thermique par l'extérieur.

par le dégel de la réserve de précaution, mais aussi par une ouverture de crédits de 86,5 millions d'euros dans la troisième loi de finances rectificative, qui a créé un dispositif de « vacances apprenantes » en lien avec plusieurs ministères, dont celui de l'éducation nationale.

Le budget prend en compte une partie des coûts induits par la crise sanitaire, même si, à l'évidence, de nouvelles ouvertures de crédits seront nécessaires en cours d'année pour les APL et probablement pour l'hébergement d'urgence. Malgré cette réserve, je vous proposerai d'adopter les crédits de la mission, pour ce qui concerne les programmes que je vous ai présentés.

Enfin, je ne peux terminer, madame la ministre, sans évoquer la situation du logement en cette fin d'année, même si cette politique est de moins en moins mise en oeuvre au travers des crédits de la mission.

perspectives de la suppression de la taxe d'habitation pour les collectivités locales, non-compensation des exonérations de taxe foncière pour les bailleurs sociaux et le logement intermédiaire. Madame la ministre, il vous faut répondre sur tous ces points, et redonner rapidement de la visibilité aux acteurs, faute de quoi nous irons droit à une crise du logement sans précédent.

Mon regret concerne l'abandon du nom « ruralité » dans les nouveaux contrats avec les territoires. Les contrats de ruralité deviennent des contrats à la relance ! Certes, nous sommes dans une période de relance qu'il nous faut réussir, et tout cela n'est affaire

le secrétaire d'État, les enjeux de la ruralité doivent être bien identifiés. Ils ne peuvent pas être dilués dans d'autres enjeux nationaux, particulièrement au moment où le secteur rural retrouve de l'intérêt et de l'attractivité pour un grand nombre de Français.

L'ensemble des crédits consacrés à la politique d'aménagement du territoire, et notamment aux politiques contractuelles, sont dispersés dans plusieurs missions, ce qui est dommageable. Pour davantage de visibilité, de cohérence et d'efficacité,

en partage le vécu de la ruralité et une connaissance fine de ses enjeux, notamment des territoires de montagne. Nous comptons sur vous pour permettre aux territoires ruraux de jouer pleinement leur rôle.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, au nom de la commission des affaires économiques, je voudrais formuler trois observations : notre déception concernant la construction neuve, notre préoccupation concernant le financement des APL et notre souhait de voir s'amplifier l'effort en faveur du Logement d'abord. Concernant la construction neuve, nous regrettons qu'elle n'ait pu trouver sa place au sein du plan de relance. Son absence même ne dit-elle pas quelque chose de l'état d'esprit du Gouvernement ? Préférer isoler l'ancien plutôt que construire pour les nouveaux ménages, n'est-ce pas un signe préoccupant pour l'avenir ? Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une double occasion manquée. Occasion manquée de prendre des mesures de relance à effet immédiat, comme la remise en cause de la réduction de loyer de solidarité,

Occasion manquée aussi de prendre des mesures structurelles comme la création d'un véritable statut du bailleur privé, qui ne doit pas être considéré comme un rentier improductif, mais comme un entrepreneur du logement. Concernant les APL, je ne partage pas les craintes de certains à propos du nouveau mode de calcul contemporain des droits, qui me paraît juste et semble avoir été sérieusement préparé.

prochaine. Peut-on vraiment compter sur le budget de l'État pour y pourvoir ? Ne doit-on pas plutôt craindre que le 1 % logement soit définitivement siphonné par le Fonds national d'aide au logement ? doit-on se préparer à un nouveau coup de Jarnac au détour de la réforme du revenu universel d'activité (RUA) dont le Premier ministre a relancé les travaux ? Enfin, je veux saluer l'effort que le Gouvernement a réalisé l'an passé et qu'il va poursuivre en 2021 pour mettre les dispositifs d'hébergement et de logement accompagné à la hauteur de la crise sanitaire que nous traversons et des changements qu'elle implique. Le « quoi qu'il en coûte » trouve ici une belle et humaine illustration. Il convient de le souligner et de renouveler notre reconnaissance aux personnels du secteur. Dans son rapport sur le plan de relance, la commission des affaires économiques avait demandé l'accélération de la transformation

sur la part du plan de relance consacrée aux quartiers populaires, sur l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et enfin sur la vision qui doit animer cette politique. les maires des quartiers populaires ont lancé un appel au secours au Président de la République, en raison de la dégradation dramatique de la situation dans leurs communes : surmortalité liée à la covid-19, augmentation des demandes de RSA, explosion des aides alimentaires, chômage galopant

Deux ans plus tard, elle reste lettre morte et, au gouvernement, personne ne sait même plus de quoi il s'agit. Autre exemple, dans son discours prononcé aux Mureaux, le 2 octobre dernier,

Cette mobilisation a permis d'ouvrir 35 000 places d'hébergement temporaire au plus fort de la crise, de déployer des équipes mobiles sanitaires et de distribuer des chèques-services à près de 90 000 personnes. Cette situation exceptionnelle, qui a porté le parc d'hébergement à 180 000 places, a fait naître des besoins de financement considérables pour le programme 177, dont les crédits avaient déjà augmenté de 45 % en cinq ans, pour atteindre 2,1 milliards d'euros, en 2019. Les crédits ouverts cette année s'élèvent à 2,44 milliards d'euros, alors que la LFI pour 2020 n'avait prévu qu'une enveloppe de 1,99 milliard Si les efforts de budgétisation pour 2021 sont significatifs, des incertitudes demeurent quant au niveau de crédits qui sera nécessaire pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Dans ce contexte, la politique de l'hébergement et de l'insertion vers le logement doit répondre à trois exigences. La première sera de satisfaire les demandes d'hébergement et d'accompagnement de nos concitoyens, qui risquent d'être

La deuxième exigence est de poursuivre activement le plan du logement adapté qui a été freiné par la crise. À ce stade, l'objectif de créer en cinq ans 10 000 places en pension de famille et 40 000 places en intermédiation locative risque de ne pas être atteint. Saluons cependant la hausse de 16 à 18 euros du financement par place en pension de famille. Il convient de poursuivre ce soutien, notamment en faveur des résidences sociales, afin de renforcer l'insertion vers le logement et de limiter le recours aux dispositifs d'urgence. Enfin, de manière les chantiers de rationalisation et de gouvernance doivent être menés à terme, ce qui prendra du temps. Les acteurs du monde associatif ont un rôle à jouer dans le cadre d'un plan de cohésion sociale, devenu non seulement une exigence, mais aussi une priorité.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous indique d'emblée que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable à l'adoption des crédits aux politiques des territoires des programmes 112 et 162. Elle a toutefois formulé plusieurs réserves et je vous ferai part de deux observations et deux questions. D'abord, et je m'en réjouis, le budget consacré aux projets et aux politiques de nos territoires est en hausse, cette année, grâce aux crédits inscrits dans la mission « Plan de relance ». Cet effort est suffisamment rare pour être relevé, car les crédits du programme 112 ne cessent de diminuer depuis plusieurs années. C'est pourquoi je salue le renforcement des moyens du programme France Services, même si des progrès restent à faire pour rapprocher l'offre de services de nos concitoyens. Le critère de distance, fixé à trente

je salue le doublement à 20 millions d'euros des crédits d'ingénierie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, pour sa deuxième année d'existence. Cette enveloppe sera enrichie de la trésorerie restante sur la ligne « Ingénierie » du budget pour 2020, ainsi que d'un apport de 9 millions d'euros de la Banque des territoires pour le programme « Petites villes de demain ». Elle devrait permettre à l'agence d'intervenir efficacement cette année. À cet égard, je souhaite vous interroger, monsieur le secrétaire d'État : pouvons-nous espérer que les moyens de l'ANCT consacrés à l'ingénierie de projets suivent une trajectoire d'augmentation pour les prochains exercices ?

Si le programme Territoires d'industrie prend le relais, son périmètre d'intervention géographique me semble trop restreint à ce jour : il faudra aller au-delà des 148 territoires déjà ciblés. Surtout, je voudrais insister- comme mes collègues ont déjà pu le faire -sur le manque de lisibilité de ce projet de loi de finances pour 2021. Trop nombreux sont les crédits inscrits dans la mission « Plan de relance », alors qu'ils ont vocation à financer des actions entrant dans le périmètre des programmes budgétaires de droit commun, comme les programmes 112 et 162. Cela introduit une confusion qui n'est pas souhaitable. Je rappelle en outre qu'en mettant à part le plan de relance les crédits du programme 112 baissent de 15 % en autorisations d'engagement et de 4 % en crédits de paiement.

seront-ils reportés sur le programme 112, annulés ou redistribués ? La parole

politique aujourd'hui pilotée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont nous examinons les crédits aujourd'hui. Je rappelle que le plan de relance consacrera 240 millions d'euros au plan France Très haut débit, afin d'assurer la couverture intégrale du territoire en fibre optique d'ici à 2025, portant à 550 millions d'euros les crédits supplémentaires alloués au déploiement des réseaux fixes. d'un motif de satisfaction majeur pour notre assemblée qui, depuis plusieurs années, a engagé un combat pour assurer la couverture numérique des territoires. Ces crédits devront maintenant être déployés sous l'autorité de l'ANCT et selon des modalités fixées par un cahier des charges, qui déterminera les conditions de financement des réseaux d'initiative publique par l'État et influencera, en conséquence, les taux de cofinancement du secteur privé et des collectivités territoriales. Une nouvelle version de ce cahier des charges sera très prochainement publiée. Il faut espérer qu'elle se traduise par une augmentation effective du soutien de l'État dans les territoires, à accompagner le déploiement de la fibre en zone d'initiative publique, mais également à financer les raccordements dits « complexes » en zone publique ou privée. Il s'agira pour nous d'un point de vigilance Je rappelle que l'ANCT joue également un rôle pilote dans la mise en oeuvre du « New Deal mobile », accord conclu en 2018 entre l'État et les opérateurs, visant à améliorer la couverture mobile et à résorber les zones blanches. blanches. Ce programme de déploiement des réseaux mobiles ne fait pas l'objet d'un soutien budgétaire spécifique, l'État ayant renoncé au produit des redevances, estimé à 3 milliards d'euros, en contrepartie de la souscription d'engagements contraignants Plus de deux ans après le lancement du « New Deal », le bilan est plutôt positif. Concernant le dispositif de couverture ciblée pour lutter contre les zones blanches, plus de 90 % des 445 sites identifiés dans le premier arrêté ont été livrés dans les temps. Les retards résiduels devront être dûment justifiés, mais on peut se féliciter globalement de la dynamique actuelle. Concernant l'objectif de généralisation de la 4G sur les sites existants, l'objectif devrait également être tenu. Au total, 96 % de la population est aujourd'hui desservie en 4G par au moins un opérateur, et 76 % par les quatre grands opérateurs. Sur ce volet relatif aux infrastructures, le travail mené sous l'autorité de l'ANCT avance donc à un bon rythme. Notre commission maintiendra sa vigilance pour s'assurer de la poursuite de cette dynamique et, surtout, veillera à ce que les engagements pris au service de la cohésion des territoires Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

Le confinement a également mis en évidence des inégalités insupportables au regard des conditions de logement. Enfin, la crise sociale a accru les problèmes de pouvoir d'achat des Français modestes, des classes moyennes et, surtout, aggravé

Le logement coûte trop cher aux Français et nécessiterait une politique volontariste de régulation des prix, tant des loyers que du foncier. Mais il n'en est rien

Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, et bien avant la crise du covid, la pauvreté s'est accrue en France. Les études montrent que la baisse des APL en constitue l'une des causes majeures. Si les Français n'ont pas vu les effets du ruissellement, beaucoup ont subi une douche froide ! Notre groupe a déposé une proposition de loi sur la revalorisation des APL et la suppression du mois de carence.

en particulier avec la réforme de la contemporanéisation des APL, dont on peut discuter le principe- qui pourrait paraître juste -, mais dont les conditions de mise en oeuvre ont constitué un grave recul pour bon nombre de nos concitoyens. L'État fera une économie de 750 millions d'euros, même si l'on prend en compte la dégradation des ressources liée à la crise. Ces 750 millions d'euros seront prélevés sur les familles modestes : c'est une véritable injustice

la France a massivement besoin de logements sociaux en locatif et en accession. Zéro euro pour l'aide à la pierre destinée au logement social, d'un côté ; 1,2 milliard d'euros inscrits au budget au titre des aides fiscales de type Pinel,

La chute des aides à la pierre pour les HLM non seulement obère la construction, mais conduit à fixer des loyers de sortie trop élevés au regard des ressources de nos concitoyens. Il faudrait baisser le taux de TVA à 5,5 %, supprimer la RLS et créer une prime pour l'accession vraiment sociale tout cela, hélas, n'est pas dans ce budget. C'est pourquoi nous défendrons des amendements en ce sens. Enfin, la situation exigerait une mobilisation sans précédent de l'État pour la politique de la ville et en direction des quartiers populaires, que la crise percute de plein fouet, mais qui étaient déjà en terrible difficulté et trop négligés auparavant. Ils ont impérativement besoin d'investissements publics massifs humains, éducatifs, de soutien à l'insertion, à l'emploi, aux initiatives associatives et citoyennes. Ils ont besoin d'un retour des services publics et d'un en matière de renouvellement urbain. C'est ce que demandent les maires à travers l'appel qu'ils ont lancé il y a peu. Nous soutenons pleinement leurs revendications. Monsieur le secrétaire d'État, madame la ministre, ils doivent être entendus : les promesses qui leur sont faites doivent être vraiment tenues, en particulier le milliard d'euros du plan de relance ; et surtout, l'argent doit parvenir réellement et vite sur le terrain. Cela changera

à l'impératif républicain, qui exigerait que la Nation se mobilise fortement, à la fois pour le droit au logement et pour une politique de la ville ambitieuse. Le groupe CRCE ne votera donc pas les crédits

Nous les évoquions depuis longtemps, la pandémie de la covid-19 les a exacerbés. La violence de la crise nous a obligés, à plusieurs reprises au cours de l'année 2020 sous la forme de projets de loi de finances rectificative successifs, à consolider certaines politiques et certains programmes, qui touchent à la mission « Cohésion des territoires ». Je pense bien sûr aux politiques ciblant les plus vulnérables, qui sont durement touchés par les conséquences sanitaires et économiques de la crise. Je tiens à saluer les efforts que le Gouvernement a déployés ces derniers mois, particulièrement en matière d'hébergement d'urgence. Le groupe Les Indépendants est favorable à l'adoption des crédits de la mission à plusieurs titres. Quatre dossiers que nous sommes nombreux à partager dans cet hémicycle me semblent aller dans le bon sens en matière de cohésion de nos territoires. Le premier est celui de la politique de la ville, qui favorise des programmes de rénovation dans de nombreuses communes, qui permet d'améliorer le bien-être de familles entières, de répondre aux difficultés des populations jeunes et souvent pauvres, de faire revivre des quartiers entiers. Le deuxième est celui de la prime à l'aménagement du territoire. Ce dispositif a prouvé son importance pour le dynamisme de nos territoires et celui de leur tissu économique. Sa prorogation est souhaitable. troisième concerne les zones de revitalisation rurale qui voient leur existence prorogée jusqu'en 2022 : c'est un point à saluer, de même que la reconduction de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), de la

ont été marqués par la complexité de la crise et l'arrivée de nouveaux élus qui, eux aussi, ont été absorbés par la gestion de la pandémie. Je salue la hausse des moyens consacrés à l'ANCT, particulièrement les crédits destinés à l'ingénierie des collectivités territoriales, qui sont multipliés par deux. L'Agence doit réussir, surtout dans la ruralité : nous resterons vigilants à ce qu'elle soit toujours dotée de moyens suffisants pour exercer ses missions. Je souhaite terminer en soulevant deux points de vigilance. D'abord, mon groupe a, à plusieurs reprises, alerté sur le manque de cohérence et d'accessibilité de certains programmes et des moyens complémentaires figurant dans

notamment dans le secteur de la santé. L'an dernier, nous avions exprimé des préoccupations quant à leur financement ; aujourd'hui, je veux rappeler le caractère primordial des CPER pour les projets prioritaires des collectivités territoriales.

La fracture numérique entre les territoires est immense ; les zones blanches sont encore, comme le très faible débit, monnaie courante ; on parle beaucoup de la 5G, mais il faut rappeler que certains territoires n'ont tout simplement pas accès au réseau : c'est une source d'inégalités profondes, et il y a urgence dans ce domaine.

Je pense à nos jeunes, dont l'éducation se poursuit en partie grâce à l'accès au numérique. Il en va de même pour nos commerces dont la numérisation s'est accélérée. Les crédits qui sont alloués au plan France Très haut débit semblent emprunter un chemin satisfaisant. Nous devons accélérer collectivement cette transition. Au total, la mission reflète plusieurs intentions : une plus grande implication des collectivités territoriales, une réponse davantage différenciée selon les enjeux de chaque territoire, une plus grande cohésion dans leur aménagement. L'ensemble de ces ambitions s'inscrit, enfin, dans le cadre de la transition écologique, ce qui nous paraît aller dans la bonne direction.

Cette crise implique donc un renforcement en urgence de plusieurs dispositifs de politique publique pour soutenir les plus fragiles, en intégrant ces nouveaux publics, étudiants, commerçants et entrepreneurs individuels, qui ont basculé dans la précarité. Il se trouve, madame la ministre, que nous nous sommes réunis à Nantes pour discuter de ces sujets. Les témoignages qui remontent des associations sont extrêmement inquiétants à cet égard. Dans ce contexte, la mission « Cohésion des territoires », qui regroupe l'action publique en matière d'hébergement, de parcours vers le logement et d'insertion des personnes vulnérables ou d'amélioration de l'habitat, est un axe fort du projet de loi de finances et mérite une attention toute particulière. Or l'effort budgétaire fourni par le Gouvernement ne nous semble pas à la hauteur de nombre de ces enjeux. Tout d'abord, la politique du logement a été mise à mal ces dernières années. Les crédits des APL ont fortement diminué depuis 2017, alors que l'accès au logement implique que l'on prenne des mesures très fortes. Nous avons donc déposé une série d'amendements tendant à financer l'accompagnement social dans le cadre du plan quinquennal pour le Logement d'abord, ou à renforcer concrètement- c'est une demande précise -les capacités d'accueil des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences. Avec le confinement, nous le savons, les violences conjugales ont en effet beaucoup augmenté.

Dans un rapport publié la semaine dernière, le Haut Conseil pour le climat constate un retard de la France par rapport à ses voisins européens dans ce domaine pourtant indispensable à la transition écologique. Il recommande notamment de mieux dépenser l'argent public et de le flécher vers des rénovations en profondeur.

fameux nouveaux contrats de relance et de transition écologique, qui restent encore assez mal définis. J'ai d'ailleurs trouvé notre collègue Bernard Delcros très optimiste sur ce point. Il a peut-être des informations dont je ne dispose

à énergie positive, ou les contrats de transition écologique (CTE). Les collectivités ont besoin de stabilité et de visibilité. Il aurait suffi de contractualiser sur le fondement du plan climat-air-énergie territorial

ce même programme 112 les crédits de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui a maintenant un an d'existence. En tant que guichet unique chargé de l'accompagnement en ingénierie des élus, notamment pour le déploiement de différents programmes nationaux, l'Agence demande évidemment des moyens humains importants.

Pour déployer le plan de relance sur le terrain, le compte n'y est donc pas. Il importe de donner à l'ANCT des moyens humains et budgétaires à la hauteur des enjeux auxquels la population et les collectivités territoriales sont confrontées, à la hauteur de leurs attentes. Nous avons donc déposé un amendement ayant pour objet de les augmenter. Concernant la politique de la ville, nous devons aussi amplifier nos actions en faveur de l'emploi, de l'éducation prioritaire et du renouvellement urbain, comme l'a dit Marie-Noëlle Lienemann. Sur ce dernier point, la dotation de l'État est en deçà de la trajectoire annoncée et les incertitudes liées à l'avenir du groupe Action Logement, financeur majeur, font peser de vraies craintes sur l'avenir. Je n'ai pas l'habitude de citer le rapporteur Dallier dans le texte tous les jours, ... Tout arrive ! Vous avez tort de ne

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons actuellement nous montre combien la cohésion des territoires est essentielle dans notre pays. Elle requiert ce soir toute notre attention, dans la chambre des territoires. Au coeur des préoccupations des Français, la mission « Cohésion des territoires » est composée de six programmes et regroupe plusieurs politiques intégratrices : le logement, l'hébergement et l'insertion des personnes vulnérables, l'aménagement des territoires et la rénovation énergétique. Pour l'année 2021, les crédits de cette mission s'élèvent à 16 milliards d'euros, soit une hausse de 5,3 % par rapport à 2020. Ils sont à la hauteur des objectifs nous nous sommes fixés depuis trois ans, afin d'accompagner les territoires dans leur diversité, réduire les inégalités, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens où qu'ils habitent. En cinq minutes, je ne pourrai pas détailler l'ensemble de ces crédits, mais permettez-moi, mes chers collègues, d'insister sur les trois principaux axes qui me semblent faire la force de cette mission. porte sur l'hébergement, l'insertion des personnes vulnérables et le logement. Dans le contexte de la crise sanitaire qui marque cette année 2020, les actions en faveur du logement, de l'hébergement et de l'insertion des personnes vulnérables ont été fortes. de la mise à l'abri et l'impérieuse nécessité de protéger les personnes à la rue, vivant dans des squats ou des campements, du risque de contamination, environ 30 000 places d'hébergement ont pu être ouvertes. Les crédits de cette mission contribuent également à assurer un meilleur repérage des personnes hébergées ou à la rue, qui peuvent accéder à un logement. Cela passe par un effort budgétaire significatif pour les maraudes, soit 12 millions d'euros supplémentaires pour consolider les réponses apportées aux personnes en situation d'exclusion, dont 4 millions d'euros pour les accueils de jour et 8 millions d'euros pour le renfort des services intégrés de l'accueil et de l'orientation. Cela passe également par la création de 1 000 places d'hébergement supplémentaires destinées aux femmes des victimes de violences parmi les 14 000 nouvelles places d'hébergement prévues en 2021. Ensuite, 80 % des crédits de la mission sont concentrés sur deux postes principaux. Il y a, d'une part, l'aide dite « à la personne », ciblée sur les ménages aux ressources les plus modestes, qui constitue le principal poste budgétaire de la politique du logement. L'ensemble des prestations devraient s'élever à 15,7 milliards d'euros en 2021, dont 78 % du montant total des aides personnalisées au logement le Fonds national d'aide au logement, le reste du financement étant principalement assuré par les cotisations des employeurs. Il y a, d'autre part, l'accès au logement décent. décent. Le programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat », qui regroupe les crédits relatifs à la construction, à l'urbanisme et à l'aménagement, est l'un des outils majeurs pour la mise en oeuvre opérationnelle des politiques liées au logement, avec un budget de 528 millions d'euros. Ces crédits sont complétés par les crédits de la mission « Plan de relance » consacrés à ces politiques, qui s'élèvent à 7,2 milliards d'euros.

Intervenant dans 1 514 quartiers prioritaires, qui correspondent aux principales concentrations urbaines de la pauvreté en métropole et en outre-mer, la politique de la ville relève du droit commun et bénéficie d'un budget de 515 millions d'euros,

par rapport aux précédents quinquennats. Les moyens financiers affectés aux quartiers prioritaires de la ville continueront d'augmenter, avec la pérennisation des 1 514 nouveaux postes d'adultes-relais créés à l'été 2020 dans le cadre des opérations Quartiers d'été, le déploiement des cités de l'emploi et l'augmentation des crédits de l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi à hauteur de 32 millions d'euros. Le nouveau programme de rénovation urbaine sera également amplifié et doté de 10 milliards d'euros, afin de soutenir 480 projets et de financer 44 associations qui contribuent à des actions innovantes à travers l'appel à manifestation d'intérêt « Tremplin Asso ». Par ailleurs, nous pouvons saluer l'augmentation de 17 millions d'euros du programme consacré aux cités éducatives qui, pour rappel, constituent une démarche collective permettant à l'ensemble des acteurs et des lieux éducatifs de travailler en synergie dès la maternelle jusqu'à l'insertion professionnelle des jeunes adultes pour garantir la réussite scolaire de chaque enfant. C'est aussi par l'éducation que nous renforçons l'égalité des chances. Le troisième et dernier axe est le soutien aux territoires et à la coordination territoriale. En 2021, le soutien aux territoires s'appuiera largement sur l'accélération de l'inclusion numérique et du plan France France Très haut débit. Ces actions seront mises en oeuvre, notamment dans le cadre de la nouvelle génération des contrats de plan État-région et des contrats de plan interrégionaux État-région 2021-2027, et par le biais de l'ANCT, dans une logique de proximité, afin d'appréhender au mieux les besoins de chaque territoire. D'autres programmes spécifiques viendront accompagner les grandes transformations territoriales. Je pense aux programmes « France Services », « Territoires d'industrie », « Nouveaux lieux, nouveaux liens », « Action coeur de ville », « Petites villes de demain », ou encore à l'« agenda rural », un sujet auquel je suis, comme beaucoup d'entre vous, vous, très sensible. Monsieur le secrétaire d'État, je vous rappelle que le Gouvernement avait retenu 173 propositions : vous nous direz où nous en sommes de l'application de ces mesures. Enfin, en matière de coordination territoriale, la mission comporte des actions territorialisées, qui répondent à des enjeux divers témoignent de l'engagement de l'État sur son territoire. Logement, politique de la ville, soutien et coordination entre territoires, tels sont les points forts de cette mission. C'est pourquoi le groupe RDPI votera les crédits de la mission « Cohésion des territoires

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la pandémie du covid-19 qui nous touche depuis près d'un an a, et aura, des conséquences sanitaires, sociales, économiques que nous devrons collectivement affronter. Le montant total de cette mission s'élève à 15,91 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 15,99 milliards d'euros en crédits de paiement, en légère augmentation par rapport au montant des crédits attribués en 2020. Nous avons souhaité, en cette année si particulière, faire porter l'effort sur quelques secteurs plus saillants. Ainsi, nous vous proposons de conforter les crédits destinés aux hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violence, ainsi que les APL accession, mais aussi de nous associer à des mesures complémentaires de soutien pour nos commerces de proximité. Nous n'oublions pas pour autant les conséquences territoriales de cette pandémie, qui toucheront davantage des territoires déjà fragilisés et visés, à ce titre, par des politiques de cohésion. Aujourd'hui, nos élus s'inquiètent du fait que leur projet de dynamisation de leur commune soit durablement marqué par de possibles faillites de commerçants, l'annulation de fêtes ou de festivals. Et j'aurai, à cet égard, une pensée particulière pour les élus de moyenne montagne : la neige ne sera pas

Ces abondements supplémentaires sont évidemment les bienvenus, si tant est que ces aides de relance économique soient bien accessibles à tous, visibles et fléchées. Nous sommes aussi vigilants à ce qu'elles ne se substituent pas à des engagements pérennes menés depuis des années. La mise en oeuvre de la deuxième génération de l'agenda rural, le désenclavement des territoires et, en particulier, la pérennité des crédits mobilité qui viendront abonder les CPER pour les nouveaux contrats de transition écologique et le plan France Très haut débit à destination de la ruralité constituent la colonne vertébrale de nos politiques d'aménagement du territoire, qui ne devront en aucun cas être sacrifiées. Faute de quoi, l'ensemble des crédits de la relance ou de cohésion perdront de leur efficacité. Or les abondements prévus au programme 112 nous paraissent fragiles. Plus que jamais, en effet, nous avons besoin d'outils administratifs opérationnels, simples, présents physiquement dans nos territoires, au service de nos projets locaux. L'Agence nationale de la cohésion des territoires, née sur l'initiative du groupe du RDSE, entrera en 2021 dans sa première véritable année d'existence. Lors de sa communication d'étape, en juillet 2020, devant la délégation aux collectivités territoriales, notre ancienne collègue Josiane Costes avait rappelé quelle était notre première préoccupation : il s'agit bien d'assurer « l'appui en ingénierie et sur mesure à des projets locaux développer du bas vers le haut, et non du haut vers le bas ». Or les remontées que nous avons des comités locaux de cohésion territoriale confirment nos craintes initiales que l'agence ne se dilue dans ses multiples responsabilités nationales. Nous devons infléchir cette tendance. Aussi, mes chers collègues, nous proposons à votre vote plusieurs amendements pour conforter ses missions directes d'ingénierie territoriale. Certes, l'ANCT bénéficiera de 20 millions d'euros supplémentaires sur ces missions,

qui, en 2021, devront remettre l'ouvrage sur le métier, dans des circonstances très difficiles, pour reconstruire une vie locale avec le virus. Plus que jamais, mes chers collègues, faisons confiance à l'intelligence territoriale ! La parole

indiqué mon collègue Olivier Henno, nous saluons les mesures exceptionnelles qui ont été prises dans le secteur de l'hébergement depuis le début de la crise, afin de lutter contre l'épidémie et de protéger les populations les plus fragilisées : accroissement des capacités d'hébergement d'urgence, mise à l'abri des personnes, tout en diminuant la densité d'occupation des structures pour respecter les consignes sanitaires. Ce sont 35 000 places exceptionnelles qui ont été ouvertes, dont 14 000 seront pérennisées d'ici à 2021. Si l'on peut se féliciter de l'engagement du Gouvernement en faveur de l'hébergement d'urgence, des efforts importants sont également réalisés pour la rénovation énergétique des bâtiments et du logement, le plan de relance, qui consacre 6,3 milliards d'euros d'autorisations d'engagement à la rénovation énergétique sur la période 2021-2022. C'est nécessaire quand on sait que le phénomène de précarité énergétique touche près de 5 millions de ménages.

il est regrettable qu'aucune mesure ne vienne soutenir la construction, car c'est un véritable levier de croissance : « 100 000 logements construits équivalent à 200 000 emplois préservés ou créés Le Gouvernement a fait un premier pas à l'Assemblée nationale, avec la prorogation du dispositif Pinel et du prêt à taux zéro (PTZ). Avec des dispositions élargies, ces propositions pourraient permettre de soutenir la filière du bâtiment et de l'artisanat, et ainsi d'engager une dynamique positive pour la relance de notre pays. de notre pays. La crise, évidemment, impactera aussi le monde du logement social, dont les difficultés étaient déjà connues. Les bailleurs sociaux, fragilisés depuis 2018 par la réduction de loyer de solidarité voient leurs problématiques se renforcer-

côté, madame la ministre, vous nous avez aidés, en signifiant que le Gouvernement ne procéderait pas par ordonnance pour réformer le groupe Action Logement.

Représentant 18 % des logements sociaux en France, Action Logement aura assuré plus de 40 % de la production en 2020 ! Que serait la construction neuve sans Action Logement ? Le groupe apporte 1,4 milliard d'euros d'aides directes aux bailleurs sociaux,

aux avant-postes de la crise sanitaire et économique, témoins de la détresse des bénévoles associatifs, ayant reçu un nombre incommensurable de demandes d'urgence, ils appellent, au nom de l'égalité républicaine, à réserver 1 % du plan de relance au soutien des quartiers et des publics prioritaires.

Au-delà, la lutte contre les fractures et pour l'égalité de tous sur notre territoire passe par une meilleure politique de la ville et par de réelles stratégies d'aménagement du territoire. C'est aussi l'objet de cette mission budgétaire. Accompagner la construction et la rénovation du logement social, déployer une politique de la ville, c'est faire de l'aménagement du territoire de manière différenciée et adaptée : différenciée en fonction des problématiques locales, mais surtout adaptée aux difficultés des habitants.

au sein de la mission « Cohésion des territoires », j'aborderai le volet relatif au logement et mon collègue Serge Mérillou traitera de la politique de la ville. Le budget de 2021 pour le logement et l'hébergement est un budget de continuité, avec des crédits en faveur de l'hébergement en hausse. Mais il ne prend pas vraiment la mesure de la gravité de la situation sociale engendrée par la pandémie. La prise en compte de l'hébergement d'urgence est insuffisante et il manque des mesures fortes pour empêcher de nombreux Français de basculer dans la précarité. S'agissant du programme 109, « Aide à l'accès au logement », le PLF pour 2021 prévoit un prélèvement sur les ressources d'Action Logement de 1 milliard d'euros pour abonder le budget des aides au logement. Cette nouvelle ponction sur la trésorerie de ce partenaire de l'État risque de fragiliser l'écosystème du logement social. Or Action Logement est un acteur clé pour appréhender la période de relance, alors que la crise sanitaire que nous traversons accentue les difficultés d'accès et de maintien dans le logement et fragilise le secteur de l'immobilier et du bâtiment dans son ensemble. Dans ce contexte, le groupe doit amplifier ses financements en faveur de la production de logements sociaux,

Pour le reste du programme 109, le contexte actuel nous fait singulièrement sentir le poids des décisions successives du Gouvernement : baisse de 5 euros, gel du barème et sous-indexation des APL ; mise en place de la réduction de loyer de solidarité ; suppression de l'APL accession.

Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain continuera de soutenir le rétablissement de l'APL accession, ainsi qu'une réévaluation du montant des aides au logement. La mise en oeuvre de la réforme des APL en temps réel frappera en premier lieu les jeunes actifs à petits revenus ou ceux qui entrent dans la vie professionnelle dans un contexte économique très difficile. Nous demandons donc la mise en place d'un régime compensatoire pour les soutenir.

Le PLF pour 2021 prévoit de nouveau la suspension de l'indexation du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS, ce qui limitera le montant des économies prévues à 1,3 milliard d'euros. Certes, la mission « Plan de relance » prévoit 60 millions d'euros pour financer les travaux de rénovation énergétique et les travaux de réhabilitation lourde de logements locatifs sociaux. Pour autant, la Caisse des dépôts et consignations anticipe une baisse de production de logements sociaux de 20 % par rapport aux objectifs du pacte d'investissement. Je voudrais aussi évoquer la question de la territorialisation des politiques d'aide au logement, qui doit davantage prendre en compte les spécificités locales. L'Assemblée nationale a introduit deux articles additionnels, prolongeant le prêt à taux zéro, ainsi que le dispositif Pinel jusqu'à la fin de 2022. Toutefois, rappelons que, depuis la loi de finances pour 2018, la quotité finançable par les PTZ a été divisée par deux : elle est passée de 40 % à 20 % pour 95 % du territoire français, soit dans les zones B2 et C. Cette différence de traitement crée une inégalité territoriale. Or, c'est justement dans les zones moins tendues, où les prix d'acquisition sont encore accessibles, que le PTZ prend tout son sens. L'inégalité est aussi manifeste avec le dispositif Pinel, dont le zonage n'a pas évolué depuis 2014. Certaines collectivités en sont donc exclues, désertées par les investisseurs, alors qu'elles présentent un besoin en logements. Je terminerai enfin sur la nécessaire relance de la construction. Le 12 novembre, l'État, les professionnels et les associations d'élus locaux ont signé le pacte national pour la relance de la construction durable. Ce pacte tend à simplifier et accélérer les procédures d'urbanisme, pour limiter la baisse des mises en chantier en 2021, et d'accompagner l'émergence de projets durables de construction. Il appelle à une déclinaison à travers des accords locaux de coordination, pour fédérer les acteurs concernés par sa mise en oeuvre. C'est une bonne méthode. En conclusion, ce PLF contient, certes, une ambition fléchée sur le logement, avec, au sein du plan de relance, un effort important en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments. Mais concernant tous les dispositifs d'aide au logement et de soutien au pouvoir d'achat des Français les

Pour toutes ces raisons, et comme depuis trois années consécutives, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain demande au Gouvernement une réorientation de la politique du logement et rejette les crédits de la mission « Cohésion des territoires ». La parole

trois ans, c'est long ! Les habitants les plus modestes des quartiers de la politique de la ville l'ont appris à leurs dépens. Eux qui devaient être les « grands gagnants » du discours de Tourcoing de 2017, eux à qui le Gouvernement devait redonner espoir sont aujourd'hui les grands perdants de ce début de quinquennat. Les conclusions du rapport de Jean-Louis Borloo offraient pourtant des perspectives intéressantes pour ces quartiers délaissés par la République. Deux ans après, où sont les actes ? Une fois de plus, le Gouvernement a fait ce qu'il sait faire le mieux : communiquer ! Très bien ! Madame la ministre, je ne ferai pas de procès en inaction. Je le reconnais, quand il s'agit de favoriser les plus riches, votre gouvernement répond présent L'accroissement des inégalités depuis l'arrivée du président Macron aux responsabilités le prouve. En juillet 2018, pour renouer avec les élus locaux de la politique de la ville, le Gouvernement annonçait vouloir garantir les mêmes droits aux habitants de ces quartiers, favoriser l'émancipation et « faire République ». Alors, certes, vous avez sanctuarisé les crédits, mais c'est insuffisant. Le bilan de ces trois dernières années est vide : vide d'ambition pour les quartiers, vide de souffle, vide d'actions concrètes pour les habitants ... laissant place, souvent, à un sentiment d'abandon, un sentiment de « non-assistance à territoire en danger Madame la ministre, il y a urgence ! Je vous le demande : écoutez les élus de terrain ! Le 14 novembre dernier, ils ont été plus de 150 à interpeller le Président de la République. Dans un courrier, ils exprimaient ainsi leur désarroi face à la politique d'abandon des quartiers menée par votre gouvernement : « Il serait Il serait irresponsable de nier que la haine et le repli sur soi prospèrent à mesure que la rupture sociale et la pauvreté augmentent. Ces quartiers subissent de plein fouet les conséquences économiques, sociales et sanitaires de la crise. Or, paradoxalement, la politique de la ville est l'angle mort du plan de relance. Madame la ministre, il nous faut renouer avec ce qui fait la grandeur de notre nation. Solidarité et fraternité doivent être les maîtres mots de la politique de relance. C'est dans cette logique que le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et moi-même proposons d'agir suivant trois axes. nous devons soutenir la mobilisation des acteurs et redonner confiance et espoir aux habitants. Le plan de relance doit être l'occasion de redonner vie à la République dans les quartiers de la politique de la ville, de restaurer la cohésion dans notre pays. Nous avons proposé dans le cadre de la mission « Plan de relance », la création d'un Conseil national des solutions composé d'élus, d'associatifs, de fonctionnaires, d'entrepreneurs et d'universitaires bénévoles. Nous n'avons pas été entendus. Ce conseil aurait vocation à identifier, promouvoir et évaluer les solutions qui fonctionnent sur le terrain en matière d'emploi, de citoyenneté, d'éducation, de sécurité, de mobilité ou encore de logement. Il aurait également comme première mission de mettre en place des collectifs pour l'emploi et la formation dans les cent villes les plus pauvres de France. Nous devons ensuite envoyer un signal fort à la jeunesse. Le PLF pour 2021 prévoit la création de 20 cités de l'emploi au bénéfice des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Nous tenons beaucoup, madame la ministre, à la création de 80 cités de l'emploi supplémentaires, pour un montant de 9 millions d'euros voté dans le cadre du plan de relance. Nous tenons également beaucoup aux propositions de la rapporteure pour avis Viviane Artigalas en faveur d'un doublement des moyens du programme de réussite éducative et de la création de 40 cités éducatives supplémentaires. Ces propositions pour la jeunesse de ces quartiers répondent à une attente forte des maires des quartiers populaires. Enfin, nous devons faire de l'ANRU un acteur de la relance dans les quartiers de la politique de la ville. À cet égard, nous nous félicitons de l'adoption par le Sénat, la semaine dernière, de l'amendement de Viviane Artigalas, tendant à augmenter de 100 millions d'euros l'investissement de l'État dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Madame la ministre, nous devons agir, et agir vite. Il y a urgence

avant tout, je veux remercier nos rapporteurs de la politique des territoires, Bernard Delcros et Louis-Jean de Nicolaÿ, pour leur travail. Sachez, mes chers collègues, que vous avez beaucoup de chance En effet, il aura fallu attendre la crise des « gilets jaunes » et la crise sanitaire pour se rendre compte de la nécessité de ne pas oublier les territoires, en particulier les territoires ruraux, qui jouent un rôle essentiel dans la cohésion économique et sociale.

l'évolution des crédits destinés à l'ingénierie de 10 millions d'euros à 20 millions d'euros en 2021. Nous nous réjouissons également de la naissance d'un nouvel outil de contractualisation avec les territoires, le programme « Petites villes de demain ».

portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs. À cette occasion, nous avions milité pour que l'on prête une attention particulière aux plus petites villes, qui étaient jusqu'alors les « oubliées » de l'aménagement du territoire.

l'ouverture du chantier destiné à réformer les critères et les mécanismes financiers associés aux ZRR. Sachez que le Sénat, maison des territoires, sera plus que jamais vigilant sur ce sujet. En effet, nous tenons aux ZRR. Plus encore, nous pensons qu'elles peuvent et doivent être un levier essentiel pour une politique de relocalisation. cette relocalisation ne se fera pas là où c'est déjà mouillé, sans que jamais le ruissellement arrive jusqu'aux territoires ruraux.

La première inquiétude porte sur l'avenir de la prime d'aménagement du territoire, qui se réduit comme peau de chagrin. J'espère que les amendements visant à rehausser les crédits de la PAT seront adoptés. La seconde interrogation concerne la distribution des crédits de l'ANCT. L'absence de lisibilité nous inquiète : à quels territoires profitera la hausse de 10 millions d'euros ? Est-ce aux petites communes, aux intercommunalités ou encore aux départements ?

d'une transversalité ministérielle qui complexifie la lecture de la mission « Cohésion des territoires ». On reproche souvent aux élus de ne pas assez utiliser les outils qui leur sont destinés : mais comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent, dans un tel labyrinthe ? C'est pourquoi je souscris à la recommandation de nos rapporteurs, qui vous demandent de rassembler tous les crédits, et principalement ceux alloués aux politiques contractuelles, au sein d'une même mission. Malgré tout, comme l'a dit mon collègue Mathieu Darnaud, les élus du groupe Les Républicains voteront les

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire a rappelé les difficultés, mais aussi les atouts de nos territoires, notamment en zone rurale. Je veux les saluer, car ils portent en eux les solutions de demain : ce sont des emplois qui peuvent être créés. À cet égard, je regrette les faibles dotations des programmes 112, « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », et 162, « Interventions territoriales de l'État ». Certes, ces programmes représentent 200 millions d'euros, mais, sur un total de 8 milliards d'euros consacrés à l'aménagement du territoire, c'est bien peu Concernant le programme 112, la baisse de 32 millions d'euros en autorisations d'engagement et de 13 millions d'euros en crédits de paiement par rapport à 2020 est significative. On invoque le plan de relance, qui absorberait un grand nombre de crédits. L'explication est recevable, mais elle ne saurait masquer une baisse de crédits de paiement pour certains dispositifs. Les députés de la majorité à l'Assemblée nationale l'ont Certains dispositifs subissent cette baisse et sont voués à disparaître, comme la prime d'aménagement du territoire, qui a bénéficié aux PME et maintenu des emplois. Elle doit être prolongée, à l'instar des zones de revitalisation rurale : la date butoir du 31 décembre 2020 est un couperet brutal. Certes, on nous annonce l'augmentation des moyens en ingénierie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, soit plus de 9 millions d'euros, et des maisons France Services. Mais puisqu'on veut aider la ruralité, j'invoquerai le bon sens paysan : nous attendons surtout des preuves Or, à ce jour, en raison du contexte, qui a ralenti son fonctionnement, l'ANCT n'a pas été en mesure d'entrer en action. Nous n'avons pas pu dresser son bilan. Pourtant, elle est appelée à jouer un rôle, notamment dans la relance. La relocalisation productive fera figure de test. L'objectif ambitieux de création ou de maintien de 13 000 emplois dans la relocalisation territoriale sera donc regardé avec attention. Quant aux maisons France Services, nous attendons aussi de constater leur valeur ajoutée par rapport aux anciennes maisons de services au public (MSAP). Cela passe par une labellisation de la part des élus. L'objectif pour 2021 d'un taux de réalisation des démarches sans redirection de 90 % est très ambitieux : ne décevons pas les espoirs qu'il inspire. La communication intensive du Gouvernement ne doit pas déboucher sur des déceptions.

Il faudra également mesurer l'efficacité de terrain des huit actions de cette mission. Les projets doivent être appuyés, car la crise sanitaire a ralenti le déploiement de certains d'entre eux. Mais ce sont surtout les populations locales qui jugeront les résultats de ces plans. Bref, les moyens accordés sont en baisse et nous le regrettons. On peut heureusement compter sur la sagesse du Sénat pour que certains crédits alloués soient augmentés. La cohésion de nos territoires doit rester prioritaire et la crise sanitaire actuelle exige des soutiens supplémentaires, car le déconfinement risque d'être plus sensible que le confinement lui-même. Malgré notre déception, nous voterons donc les crédits de ces missions

Le 16 octobre 2017, dans mon département, l'Essonne, plus d'une centaine de maires lançaient l'appel de Grigny en faveur des quartiers populaires, après quarante ans de politiques de la ville aux résultats notoirement insuffisants- c'est un euphémisme. Le 14 novembre 2017, Emmanuel Macron prononçait le discours de Tourcoing, dans lequel il annonçait un plan de mobilisation nationale pour les quartiers populaires, confié à l'ex-ministre de la ville Jean-Louis Borloo. On connaît la suite

C'est un véritable appel au secours pour non-assistance à territoire en danger. Que s'est-il passé en trois ans ? Seules quelques mesures ont pu être engagées, portées principalement par les villes elles-mêmes.

aucune mesure ambitieuse n'a été prise pour répondre à la détresse sociale et économique des communes concernées et cette inertie se paye. Aujourd'hui, un autre virus se développe dans les quartiers et même au-delà, celui du décrochage à la politique, et ce ne sont pas des lois fumeuses sur le séparatisme qui y changeront quelque chose ! De nombreux voyants sont passés au rouge. Les demandes d'aide alimentaire explosent. Le chômage augmente dangereusement.

Au regard de cette situation alarmante, le projet de loi de finances pour 2021 affiche aujourd'hui une triste réalité : les villes et les quartiers prioritaires restent un angle mort du plan de relance. L'absence de choix est le signe patent d'un manque de vision. signe patent d'un manque de vision. L'ANRU a redémarré, mais le Gouvernement, lui, est resté au bord de la route. Force est de constater que l'ambition formulée par le Président de la République- changer le visage des quartiers d'ici à la fin du quinquennat -a fait long feu. La cohésion des territoires n'est pas une vaine politique : il s'agit de permettre à l'ensemble de nos concitoyens de vivre dans des conditions décentes. Madame la ministre, il serait grand temps d'agir, car tout cela ne pourra plus durer bien longtemps

vous le savez, le logement est au coeur des préoccupations de nos concitoyens et la crise sanitaire a montré à quel point il était important d'accompagner ce secteur pour offrir à chacun un lieu de vie décent. Pour faire face à cette crise, sanitaire autant qu'économique, des moyens substantiels sont mobilisés dans le cadre de ce projet de loi de finances, qu'il s'agisse des différents programmes budgétaires concernant le logement au sein de cette mission ou des crédits de la relance.

trois priorités animent mon action ministérielle. Premièrement, je veux mener une politique d'accès au logement plus juste et plus solidaire. En cette période de crise, le budget consacré aux aides personnalisées au logement sera doté de 500 millions d'euros supplémentaires, pour atteindre 15,7 milliards d'euros. La réforme des APL en temps réel, effective à compter du 1 janvier 2021, permettra de mieux accompagner les Français dont les revenus ont diminué en raison de la crise. Cette réforme contracyclique de justice sociale est particulièrement importante dans la période actuelle. Par ailleurs, le Gouvernement mobilise des moyens sans précédent pour favoriser l'accès au logement des personnes sans domicile fixe, qu'elles soient à la rue ou hébergées. Le projet de loi de finances pour 2021 dote ainsi le programme 177 de 2,2 milliards d'euros, soit une hausse de 209 millions d'euros par rapport à 2020. Concrètement, cet effort permettra de pérenniser 14 000 nouvelles places d'hébergement et de recruter 150 personnels supplémentaires au sein des services intégrés de l'accueil et de l'orientation dans chaque département, pour améliorer l'orientation et la prise en charge des personnes sans domicile. Dans le cadre de l'acte II de la stratégie Pauvreté, ce programme bénéficie de moyens supplémentaires qui permettront notamment d'ouvrir 1 500 places d'hébergement pour les femmes sortant de maternité et de financer vingt-cinq équipes mobiles de prévention des expulsions locatives. De plus, je confirme l'engagement du Gouvernement dans le déploiement du plan Logement d'abord. Ce projet de loi de finances donne au ministère les moyens d'une véritable accélération dans l'application de ce plan, seulement par le financement de nouveaux territoires de mise en oeuvre accélérée du plan Logement d'abord, mais aussi par le renforcement du financement des pensions de famille, avec une revalorisation très attendue du forfait journalier. Ce dernier passe de 16 à 18 euros.

dont 2 milliards d'euros pour la rénovation thermique des logements privés, 4 milliards d'euros pour les bâtiments publics, 500 millions d'euros pour la réhabilitation du parc social et 200 millions d'euros pour les PME et TPE. MaPrimeRénov'est désormais la principale aide de l'État à la rénovation énergétique pour les particuliers, en complément des certificats d'énergie. Lancé en début d'année, ce dispositif connaît déjà une forte dynamique, puisque plus de 160 000 dossiers ont été déposés à ce jour. Grâce au plan de relance, MaPrimeRénov'devient accessible à tous en 2021- propriétaires et copropriétaires, bailleurs comme occupants, avec des forfaits modulés en fonction du niveau de revenus. Nous nous fixons comme objectif pour 2021 de financer plus de 400 000 rénovations ce dispositif. L'action du Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments publics est tout aussi ambitieuse. L'appel à projets lancé pour les bâtiments de l'État est un véritable succès. De très nombreux dossiers ont été déposés, allant bien au-delà de l'enveloppe prévisionnelle de 2,7 milliards d'euros. 1,3 milliard d'euros seront affectés à la rénovation des bâtiments des collectivités, en particulier les écoles, les collèges et les lycées. Nous serons particulièrement attentifs à ce que ces rénovations soient également menées dans les quartiers de la politique de la ville et concourent à l'objectif que nous nous sommes fixé : consacrer au moins 1 % du plan de relance

sur les travaux de rénovation énergétique et les critères de l'écoprêt à taux zéro. Ces dispositions permettront d'améliorer la lisibilité et la cohérence des aides à la rénovation énergétique. enfin, je suis pleinement mobilisée en faveur de la relance de la construction neuve, qui doit être une construction durable. Vous avez raison : les chiffres de la construction en 2020 sont inquiétants et nous devons faire face à cette menace. devons soutenir la construction neuve, car nous avons besoin d'un plus grand nombre de logements ; mais il faut soutenir des opérations de construction et d'aménagement durables, qui permettent également de lutter contre l'artificialisation des sols et l'étalement urbain. Au total, 650 millions d'euros y sont consacrés dans le cadre du plan de relance. Pour mobiliser l'ensemble des acteurs autour de cette démarche, j'ai signé, le 10 novembre dernier, avec les associations de collectivités territoriales et les professionnels de la construction, un pacte pour la relance de la construction durable. Ce pacte suit deux grands axes : d'une part, simplifier et accélérer les procédures soutenir l'émergence de projets de constructions durables, qui promeuvent à la fois la qualité des logements et la sobriété foncière. Il s'agit d'un acte politique fort, qui sera décliné localement en étroite collaboration avec les élus locaux, les professionnels du bâtiment et les services de l'État. Pour donner de la visibilité, on a précisé le devenir du dispositif fiscal Pinel et du prêt à taux zéro lors de l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Le prêt à taux zéro constitue le principal dispositif de soutien à l'accession à la propriété. En cette période, le Gouvernement a choisi de privilégier sa stabilité en le prorogeant jusqu'à la fin Quant au dispositif Pinel, le Gouvernement a décidé de le proroger jusqu'en 2024 tout en organisant, à compter de 2023, le transfert d'une partie du coût du dispositif en faveur du soutien au logement locatif intermédiaire géré par les institutionnels.

pour les opérations les plus vertueuses d'un point de vue environnemental ou situées dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et respectant des critères de qualité intrinsèque des logements- je pense par exemple à la taille des pièces.

au sein de la mission d'information de la commission des affaires économiques. Le Gouvernement est fermement attaché à ce qu'une réforme soit menée et souhaite travailler dans un climat de confiance avec les partenaires sociaux.

de mener à son terme la réforme de 2016 ; optimisation de la gestion et des emplois de la PEEC, afin d'améliorer l'efficacité des interventions en faveur des salariés, des entreprises et des politiques nationales du logement et de la ville. Dans un calendrier encore plus rapproché, lié au contexte économique, nous sommes convenus avec les partenaires sociaux de conclure un avenant à la convention quinquennale. Ce document permettra de déployer plus efficacement les moyens disponibles en appui du plan de relance et de discuter de la meilleure méthode permettant de soutenir le NPNRU,

Le rôle de l'État est de réduire les fractures territoriales en apportant une réponse qui tienne compte de leurs spécificités. Il s'agit de faire vivre la promesse républicaine d'égalité, en particulier d'égalité des territoires. Cet impératif est encore plus prégnant dans le contexte inédit que nous connaissons, marqué par une crise sanitaire majeure qui amplifie certaines fractures territoriales. C'est tout le sens du budget que nous vous présentons, avec un plan de relance massif et territorialisé. C'est aussi le sens des crédits de la mission « Cohésion des territoires », en particulier des programmes 112, 147 et 162, qui portent respectivement sur l'impulsion et la coordination de la politique d'aménagement du territoire, sur la politique de la ville et sur les interventions

Certes, la lecture d'ensemble est parfois peu aisée, compte tenu de la répartition des crédits entre la mission « Plan de relance » et les missions du budget général. Vous êtes nombreux à l'avoir souligné dans vos rapports

pour garantir d'ici deux ans au moins un espace France Services par canton, y compris- je le précise -dans les quartiers de la politique de la ville. Le déploiement de France Services est une mesure forte de l'agenda rural.

de l'emploi et des transitions écologique et numérique. S'y ajoute une mesure introduite par voie d'amendement à l'Assemblée nationale, que vous avez tous saluée : la prolongation de deux ans de tous les dispositifs zonés, sans exception, en particulier les zones de revitalisation rurale. C'était un engagement du Gouvernement et nous y étions tous particulièrement attachés.

Face à l'impact économique de la crise, il y a un grand enjeu de relance de l'emploi et d'accompagnement vers l'emploi, notamment pour les plus jeunes : il y va du développement attractif de nos quartiers, principe au coeur des cités de l'emploi, que nous impulsons.

C'est une méthode innovante, plébiscitée par les acteurs de terrain- certains d'entre vous l'ont rappelé -, qui travaillent ensemble avec pour seul objectif de mieux accompagner chaque jeune, pour qu'il puisse croire en ses chances. C'est aussi une occasion de réaffirmer le rôle central de l'école comme creuset républicain par excellence de l'égalité, pas simplement face aux savoirs.

Désormais, la quasi-totalité des projets sont validés ou en voie de l'être. Des chantiers sont en cours dans 230 quartiers et 10 000 logements ont déjà fait l'objet de travaux. Voilà du très concret pour les banlieues.

afin d'améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes et de renforcer leur rôle de moteur dans leur bassin de vie ; il a lancé le programme « Petites villes de demain » à destination des villes de moins de 20 000 habitants pour conforter leur rôle de centralité, renforcer le maillage du territoire et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques et sociaux à venir- annoncé en 2019, il est en train de se mettre en place.

aux bourgs-centres et aux bourgs organisés en réseau, constituant ainsi un maillage territorial au service des populations. Il s'agit, à travers ce soutien, d'améliorer le cadre de vie des populations, de favoriser le développement de ces territoires, de renforcer leur attractivité et de disposer des moyens d'accueillir les personnes qui recherchent un nouveau

La réforme dite de la contemporanéité des aides personnalisées au logement (APL) va particulièrement toucher les jeunes de moins de vingt-cinq ans. Vous nous avez confirmé, madame la ministre, lors de votre audition par la commission des affaires économiques, que les jeunes qui vont obtenir un emploi sur le marché du travail seront plutôt,

course au premier emploi, formation, stage. Faute d'un revenu minimum de subsistance dédié à la jeunesse, les APL jouent un rôle crucial pour tous les jeunes qui tentent de conquérir leur autonomie à travers une première installation dans un logement. Notre amendement tend à mettre en place une compensation pour les jeunes de moins de vingt-cinq à faibles revenus, laquelle nécessite un abondement des crédits de 300 millions d'euros. La précarité touchant 25 % des jeunes de 18 à 25 ans, il est impératif que la réforme envisagée par le Gouvernement ne vienne pas aggraver la situation. Madame la ministre, il s'agit d'un amendement d'appel : il est demandé au Gouvernement de majorer les crédits de la mission 109 en conséquence, sans faire supporter cet effort aux programmes 135 et 177 de la mission « Cohésion des territoires ». Les quatre

moins coûteux que de financer les APL pour ces ménages restant locataires. Ce dispositif a fait ses preuves, en accompagnant environ 35 000 personnes qui sont devenues propriétaires de leur logement avec une réduction moyenne de 25 % de leurs mensualités.

de mineurs de proposer à plus d'un million d'enfants et de jeunes des activités éducatives et collectives complémentaires aux apprentissages scolaires. Grâce à ce dispositif, les centres d'accueil à caractère éducatif ont pu rouvrir cet été, ce qui était inespéré

dans les projets de loi de finances pour 2020 et 2021, seuls 25 millions d'euros et 15 millions ont respectivement été inscrits en crédits de paiement. C'est d'autant plus incompréhensible que, dans son discours des Mureaux prononcé le 2 octobre dernier, le Président de la République a annoncé « un investissement supplémentaire dans l'ANRU L'État ne tient pas ses engagements, alors même que les bailleurs et les partenaires sociaux sont au rendez-vous à travers Action Logement. On comprend dès lors toute l'amertume des maires des quartiers populaires qui, dans l'appel du 14 novembre dernier, ont dénoncé les promesses non tenues et une véritable non-assistance à des territoires en danger qui décrochent de la République.

M. Michel Savin. Cet amendement vise à augmenter de 10 millions d'euros les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de l'action n° du programme 147, « Politique de la ville ». Il vise à augmenter de 50 % les moyens du programme de réussite éducative afin d'envisager son doublement sur deux ans. Ce programme repose sur l'approche globale des difficultés rencontrées par les enfants repérés dans le cadre scolaire par une équipe pluridisciplinaire de soutien ; il concentre les moyens vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les établissements scolaires inclus dans les REP+ de l'éducation nationale. mille jeunes sont actuellement ainsi pris en charge, dont 85 % bénéficient d'un parcours personnalisé. Les principales thématiques d'action sont le soutien aux parents, la santé et l'accompagnement scolaire. Après le confinement et la reprise partielle de la scolarité qui a suivi, un grand nombre d'élèves a décroché dans les quartiers populaires. Une action de grande ampleur est donc nécessaire, comme le demandent avec insistance les maires qui ont signé l'appel du 14 novembre pour éviter le décrochage de la République dans ces territoires.

vise, d'une part, à améliorer la qualité des 1 000 places qui doivent être créées en centres d'hébergement qui accueillent et accompagnent des femmes victimes de violences, d'autre part, à permettre l'ouverture de 1 000 places supplémentaires. Le Gouvernement a annoncé pour 2021 la création de 1 000 places d'hébergement sur la base d'un coût moyen de 25

des cycles de violence qu'il faut briser et dont le déroulement est bien connu : il passe par l'escalade progressive, la violence et l'explosion, qui conduit à la mise à l'abri.

centres des villages est un enjeu majeur. Des actions pour inciter les opérations de réhabilitation, de rénovation et d'adaptation de l'habitat, ainsi que les opérations de reconversion du bâti

villages et des petites villes et sauver notre patrimoine commun. Cet amendement tend à dédier une ligne de 15 millions d'euros à une aide aux maires ruraux dans leurs démarches pour favoriser ces opérations, opérations, laquelle contribuerait en outre à soutenir les TPE et l'emploi artisanal local, ainsi que la revitalisation de ces territoires. Cette proposition s'inscrit dans l'objectif de transition écologique en milieu rural du plan de relance et viendrait en complément des dispositifs de soutien à la sauvegarde du patrimoine rural. Les deux

Nous appelons cependant à davantage de déconcentration des moyens de l'ANCT et à une meilleure présence sur le terrain pour soutenir les collectivités qui en ont le plus besoin dans l'exercice de leurs compétences. Or les moyens humains de l'Agence régressent en 2021 et les préfectures, excessivement sollicitées, ne pourront pas assurer de missions supplémentaires, ce qui ne permettra pas d'instaurer une logique de guichet unique et une culture de la qualité de service. Monsieur le secrétaire d'État, le Gouvernement doit garantir aux plus fragiles des collectivités l'accès à l'expertise et à l'ingénierie territoriale ; tel est l'objectif du présent amendement, qui tend à accroître de 10 millions d'euros les crédits de l'ANCT dédiés à l'ingénierie de projet, au plus près des territoires.

du programme 147, « Politique de la ville », pour la mise en oeuvre d'un fonds de solidarité en faveur des associations sportives impliquées dans les quartiers. Ces associations sont essentielles pour maintenir le lien social, mais sont trop souvent, malheureusement, les oubliées des politiques.

La suppression de cet outil, qui accompagne le développement économique en zone rurale, pose véritablement question sur les intentions du Gouvernement. Son maintien, pour reprendre les arguments des orateurs précédents, serait cohérent avec la prorogation des zonages qui permettent de soutenir des territoires en difficulté, notamment les zones d'aide à finalité régionale, sur lesquelles la PAT peut être attribuée. Cet amendement vise à réintroduire cette prime et doter son budget de 15 millions d'euros pour 2021. Le Président de la République avait pris l'engagement d'une présence renforcée de l'État dans les territoires et d'un rééquilibrage

avis. Par cet amendement, il s'agit de sécuriser le financement du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, qui est dédié à des personnes en détresse. Il est aujourd'hui financé par des astreintes dues par l'État au titre de la mise en oeuvre du DALO, le droit au logement opposable, mais également, cette année, par un versement de 15 millions d'euros des bailleurs sociaux. Or, pendant le confinement, les astreintes liées au DALO ont été gelées et environ un tiers de leur montant devrait manquer l'année prochaine,

: La parole est à M. Jean-Yves Roux. Le logement est un lieu, où s'exercent le plus souvent les violences conjugales. Il constitue donc une question centrale pour protéger les victimes qui restent à leur domicile avec l'auteur des violences, faute de solutions alternatives. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit la pérennisation de 1 000 places supplémentaires pour un total de 6 500 places. Or, comme le souligne le rapport d'information présenté en juillet dernier par nos collègues Arnaud Bazin et Éric Bocquet relatif au financement de la lutte contre les violences faites aux femmes, le coût des premières 1 000 places n'aurait pas été budgétisé sur le programme 177 du projet de loi de finances pour 2020. Il existerait un flou sur le nombre de places réellement disponibles pour les femmes victimes de violences, d'après les associations qui sont sur le terrain. En outre, la plupart des places d'hébergement ne sont pas spécialisées dans l'accueil des femmes victimes de violences. Par conséquent, le présent amendement vise à augmenter les crédits du programme 177 de 5 millions d'euros, afin de permettre la création de 1 000 places spécialisées.

souligne la nécessité d'engager une identification et une surveillance médicale des travailleurs agricoles de la banane, en priorité, et de mettre en oeuvre sans délai les procédures en vue de l'inscription du cancer de la prostate au tableau des maladies professionnelles. Il est à noter Il est à noter que la première partie de cette recommandation semble avoir été entendue, dans la mesure où il a été fait mention d'une telle action lors des débats préliminaires à la présentation du plan Chlordécone IV. Cela répond aux demandes répétées des syndicats et des élus. Toutefois, pour que cette promesse soit effective, il faut que son action soit immédiate et d'ampleur, car nous constatons sur le terrain que les travailleurs de la banane souffrent presque tous de pathologies qui réduisent considérablement leur espérance de vie. Nous leur devons un accompagnement à la hauteur des drames qui les touchent. m'est donnée pour indiquer que nous sommes satisfaits de la publication du décret d'application relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, même si cela a pris du temps.

potentiels englobera la problématique des cancers de la prostate comme maladie professionnelle. C'est pourquoi, malgré tout et dans l'attente de votre réponse, cet amendement prévoit que la future mission dédiée à l'identification et au suivi des travailleurs agricoles de la banane

glissement de crédits a pour seul objectif de garantir la recevabilité financière de l'amendement. Compte tenu des engagements du Président de la République, qui a fixé une ambition nouvelle aux politiques publiques conduites depuis dix ans, en affirmant le devoir de transparence vis-à-vis des populations, il paraît nécessaire, pour que les crédits du programme 135 ne soient pas impactés par l'adoption de cet amendement que le Gouvernement lève le gage. L'amendement n°

de finances pour 2021 procède à une régression de ses moyens humains. La baisse de six équivalents temps plein n'est pas cohérente avec la montée en puissance de l'agence et la nécessité de mobiliser avec efficacité les crédits du plan de relance. Par le présent amendement, qui vise à augmenter d'un peu plus d'un million d'euros, ce qui est très raisonnable, les crédits relatifs à l'ingénierie territoriale, nous souhaitons budgéter le recrutement de 21 équivalents temps plein affectés auprès des territoires ruraux. Il s'agit tout simplement de traduire le souhait du Premier ministre qui, lors de sa déclaration de politique générale du 16 juillet dernier au Sénat, a affirmé que toutes les créations d'emplois autorisées par le PLF 2021 seraient destinées, sauf exception justifiée, aux services départementaux de l'État,

de venir soutenir l'ingénierie des collectivités territoriales situées en milieu rural, afin de les aider à bénéficier des moyens prévus par le plan de relance, comme cela a été annoncé par le Gouvernement lors du deuxième comité interministériel aux ruralités.

tous bénévoles nommés pour un mandat de deux ans non renouvelables. Sa mission serait de faciliter l'essaimage des expérimentations locales qui apportent des solutions concrètes aux problématiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il aurait également un rôle de vigie, qui n'est plus assuré par le Conseil national des villes et le Conseil

En application de l'article L.O. 320 du code électoral, elle est remplacée par M. Alain Sévêque, dont le mandat de sénateur de la Manche commence le 2 décembre, à zéro heure.

je trouve l'idée extrêmement intéressante, parce que les bourgs de 700 ou 800 habitants, qui ont un véritable rôle de centralité et de pôle de services pour tout un bassin de vie, ne réclament pas le statut de petite ville. On pourrait donc imaginer, monsieur le secrétaire d'État, un grand programme

C'est vrai, madame le ministre, 50 millions d'euros, ce n'est pas rien, mais c'est aussi très peu de choses ! Certains de nos collègues l'ont très bien expliqué : ce que vous donnez d'un côté pour financer l'accession à la propriété des ménages modestes,

augmentation des crédits de 31,9 millions d'euros pour améliorer l'hébergement des femmes victimes de violences. C'est un sujet que nous avons déjà évoqué dans le cadre de ce projet de loi de finances.

de loi de finances pour 2021 sont inscrits 20 millions d'euros au programme 112 pour l'ingénierie de l'ANCT, auxquels s'ajoutent 20 millions d'euros

beaucoup plus qu'il n'a pu le faire par le passé, particulièrement en cette période de crise. Une chose est certaine, en effet : si la crise sanitaire s'arrête- souhaitons-le tous -avec le vaccin,

profonde et la plus en difficulté,

Les étudiants, les apprentis, les stagiaires, vont continuer à bénéficier de règles spécifiques pour le calcul des APL. Dans leur grande majorité, ils ne verront pas leur APL évoluer. Les étudiants salariés pourront même voir leur APL augmenter grâce à la mise en place d'un forfait étudiant.

sur l'APL accession. La loi de finances pour 2018 a prévu, c'est vrai, la mise en extinction de ce dispositif, qui était en forte décroissance en volume ces dernières années. Bien sûr, les prêts signés avant 2018 restent éligibles à l'aide, une phase transitoire, jusqu'au 1 janvier 2020, a permis de ne pas remettre en cause les projets immobiliers déjà engagés. L'État dépense néanmoins toujours plus de 2 milliards d'euros par an pour aider les ménages modestes à acheter leur résidence principale.

Le déploiement du bail réel solidaire se poursuit d'ailleurs dans le cadre de ce PLF, avec notamment l'extension de l'application du taux de TVA à 5,5 % et la possibilité donnée aux collectivités de choisir le niveau d'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties. Avis défavorable sur ces quatre amendements identiques. Quel est l'avis du Gouvernement

viennent renforcer, là où il existe, le volet éducatif des contrats de ville, qui représente 26 millions d'euros ; 100 000 enfants bénéficient d'un suivi personnalisé dans ce cadre. Ces programmes sont confortés dans ce PLF, le déploiement des cités éducatives, sur lesquelles vous avez également déposé un amendement,

de son plaidoyer en faveur de l'ANAH : effectivement, cette agence, qui est financée par le programme 135, sur lequel tous ces amendements sont gagés, a absolument besoin de maintenir ses moyens pour répondre aux questions que vous posez.

est bien pris en compte dans la stratégie santé-travail du plan Chlordécone IV, dont le projet est soumis à consultation citoyenne. Il s'agit essentiellement de dispositifs réglementaires, qui seront financés par le ministère des solidarités et de la santé et l'assurance maladie.

avec les équipes de l'éducation nationale, d'organiser ce que jadis on appelait les devoirs scolaires, l'accompagnement scolaire ou l'accompagnement des personnes pour la réussite scolaire.

dépasser l'annualité budgétaire et donner des perspectives à toutes les politiques d'accompagnement des publics fragiles dans les quartiers. On fonctionne à coups d'appels à projets et d'appels à manifestation d'intérêt,

clairement identifiée, des thématiques prioritaires et la pluriannualité, vous allez faire mourir les associations et vous n'aurez plus d'excellence dans les quartiers pour accompagner les publics les plus fragiles.

vise à rattraper la perte de pouvoir d'achat subie par les ménages les plus modestes ces trois dernières années en raison des sous-indexations répétées et de la baisse de 5 euros opérée sur les APL au début du quinquennat.

Pour compenser les pertes successives de pouvoir d'achat, il est proposé de majorer les crédits alloués aux aides à l'accès au logement de 83 millions d'euros. Au regard des regrets exprimés par le Président de la République lui-même concernant la baisse de 5 euros des APL, il apparaît nécessaire que les crédits du programme 109 soient majorés par le Gouvernement, sans faire supporter cet effort par le programme 177 de la mission « Cohésion des territoires

Il est néanmoins possible qu'un abondement supplémentaire soit nécessaire en 2021, même si c'est loin d'être certain. En effet, le FNAVDL est abondé depuis 2020 à hauteur de 15 millions d'euros par an par les bailleurs sociaux, la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), ce qui représente une hausse de plus de 50 % de ses ressources et compense largement les diminutions de recettes dues au gel des astreintes.

L'appel à manifestation d'intérêt pour le logement d'abord, lancé en 2018, a concerné vingt-trois territoires, en vue de financer des mesures d'accompagnement social des personnes les plus démunies. Madame la ministre, vous avez annoncé un second appel à manifestation d'intérêt dans le but de mobiliser une dizaine de nouvelles collectivités. C'est une excellente nouvelle, car le plan quinquennal a permis le développement de nombreuses actions pour lutter contre le sans-abrisme. Cependant, alors que Paris et Marseille ont répondu à cet appel, les crédits semblent déjà insuffisants.

Pour lutter contre le sans-abrisme, amplifions une stratégie qui a donné des résultats très positifs ! Cette coopération a besoin d'ambition ; il s'agit non pas de demander du crédit pour du crédit, mais de répondre à d'autres manifestations d'intérêt que celles de Paris et Marseille.

bénéficie aux entreprises implantées sur un territoire dont les critères incluent les problématiques insulaires, est un des outils visant à pallier le cumul des contraintes « île » et « montagne » pour la Corse

la faible démographie et les incertitudes d'approvisionnement sont autant de contraintes qui entraînent des surcoûts pour les entreprises corses. Ces différents phénomènes structurels sont décuplés par l'impact de la crise sanitaire, sans précédent, dans une île dont l'économie touristique rejaillit sur l'ensemble des secteurs économiques. Ainsi, plus que jamais, il est nécessaire de proroger les dispositifs qui avaient été créés pour compenser ces contraintes. Or, si l'objectif du dispositif de ZDP est louable au regard des données précédemment évoquées, ce dernier n'a cependant pas eu les effets escomptés sur la création d'entreprises nouvelles. En effet, peu d'entreprises l'ont utilisé, privilégiant dans leur majorité le crédit d'impôt pour investissement en Corse, non cumulable avec le C'est pourquoi il est essentiel de renforcer le dispositif, en le rendant applicable aux entreprises existantes situées en milieu rural.

Il est nécessaire de muscler le dispositif de ZDP pour stimuler davantage l'activité économique productive et amortir le choc économique. Le Gouvernement a prolongé jusqu'en 2022 le dispositif de ZDP, qui devait s'éteindre amendement vise à le prolonger de trois années supplémentaires, soit jusqu'en 2025, en excluant les activités de parahôtellerie, lorsqu'elles sont créées par des particuliers dont les revenus ne représentent pas 50 % du total des revenus du foyer déclarés au titre de l'année d'imposition. Il nous semble important que le bénéfice de ce dispositif ne puisse pas être détourné pour alimenter la spéculation immobilière. La Corse, comme le pays tout entier, traverse une grave crise sociale. Lutter contre cette gangrène est particulièrement d'actualité, afin de ne pas renforcer la précarité des habitants insulaires pour l'accès au logement.

l'avis du Gouvernement ?

effet mis en dehors de tout système intercommunal et ont résisté jusqu'au dernier moment, ce qui a provoqué des situations quelque peu aberrantes. Or les maires actuels ne sont responsables en rien de cette situation dans laquelle